La séance est reprise nous reprenons la discussion du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie de la santé, du travail des transports et de l'agriculture. Dans la discussion des articles nous sommes parvenus à l'article 26. que le 26. L'amendement 21 madame Préville. Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. L'article 26, transpose dans le code de la voirie routière la directive. Européenne, du Parlement et du Conseil du 24 février 2022 qui fixe de nouvelles règles relatives à la modulation des péages autoroutiers en fonction des émissions de CO2 des véhicules de poids lourds et à la création d'une redevance pour coûts externes liés à la pollution atmosphérique pour les poids lourds en commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, le rapporteur a souhaité préciser le tonnage minimale des véhicules utilitaires lourds qui seront concernés par ces nouvelles obligations. S'appuyant sur la directive l'amendement du rapporteur adopté en commission fixe à 3,5 tonnes la valeur minimale du poids total autorisé en charge à partir de laquelle les véhicules de transport de marchandises par route et les véhicules de transport de personnes seront taxés. Nous estimons que cette valeur minimale de tonnage exclut de fait pour le transport de marchandises par route les grands véhicules utilitaires légers. Dont le poids total autorisé et généralement situées entre 2 5 et 3, 5 tonnes. Or, comme le souligne le rapport sénatorial de Madame Nicole Bonnefoy, et de monsieur Rémy Pointereau mai 2021 de la mission d'information relatives au transport de mars 10 face aux impératifs le parc de ces véhicules utilitaires légers, n'a cessé de croître ces dernières années. Ils sont de plus en plus utilisés pour le transport de fret et concurrencent ainsi les poids lourds y compris sur les longues distances et toujours d'après le rapport d'information précités. Ils sont soumis à une réglementation plus souple que les poids lourds leur développement peut dès lors, participer à une certaine sorte de déréglementation notamment sociales et environnementales du secteur par contournement des règles qui s'appliquent uniquement aux poids lourds, le risque que certaines entreprises de transport routier puisse jouer sur les effets de seuil en développant leur flotte de véhicules utilitaires légers pour échapper ainsi à la taxe est réel pour éviter un tel risque. Nous précisons, nous, nous proposons ultra-les. Utilitaires légers de transport de marchandises en permettant d'appliquer les péages dès que le poids du véhicule est supérieur à. Jusqu'. Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, cet amendement conduit à opérer une sur-transposition de la directive Eurovignette. Les nouvelles obligations imposées par la dernière version de ses directives en matière de modulation et de majoration des péages s'applique en effet aux véhicules utilitaires lourds qui sont définis comme les véhicules ayant une masse en charge maximale techniquement admissible supérieure à 3,5 tonnes. En outre, s'agissant des véhicules utilitaires légers. L'article L 122, Thierry 4 du code de la voirie routière prévoit déjà dans les futurs contrats de concession autoroutière de mettre en place une tarification différenciée selon les niveaux d'émissions des véhicules. C'est donc un avis défavorable. Monsieur le Ministre.-- Monsieur le président, Mesdames, et messieurs les sénateurs, madame la sénatrice. Monsieur le rapporteur. Même avis pour avoir une raison qui a été indiqué très précisément par monsieur le rapporteur. Nous irions au-delà des cadres de la directive et par ailleurs dans le code de la voirie routière les vu le font l'objet les véhicules utilitaires légers font l'objet d'une réglementation particulière qui peut être modulée en fonction de la performance environnementale. Mais dans le cadre de cette directive, nous ne serions. À avoir. Un changement le seuil tels que vous le proposez donc avis défavorable également. Merci, monsieur le Ministre, Madame. Oui mais justement, ce que je proposais c'était d'être plus ambitieux que ce que propose la directive européenne, ce que nous pouvons faire bien sûr et qui serait bien sûr profitable pour la transition écologique.-- Donc je mets aux voix l'amendement 21, avec 2 à 2 avis défavorable qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient. Il n'est pas adopté l'amendement 61 du gouvernement, monsieur le ministre.-- Merci monsieur le président. Les 2 alinéas 10 et 11 ont été ajoutés, l'initiative de la Commission afin de préciser que la modulation horaire des péages et la modulation CO2 de s'opérer sans recettes supplémentaires pour la concession toutefois les précisions qui ont été mentionnés, l'article dit à La Linea dise pardon sont redondantes nous paraissent pas utile et nous aurions ici une répétition du principe qu'il serait redondante et donc nuirait à la compréhension du texte. Quant à l'alinéa 11 il est pertinent, mais sa rédaction doit être légèrement pour tenir compte de cette suppression que nous proposons de l'article 10. Ce sont ces ajustements techniques qui je crois ne change pas le fond, que le gouvernement propose avec cet amendement.-- Merci monsieur le rapporteur.-- Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Donc la commission a estimé que la modulation horaire constituait une possibilité qu'il était nécessaire d'ajouter dans la nouvelle section quatre relatives aux véhicules lourds, de marchandises et de voyageurs à choisir il se d'ailleurs sans doute plus opportun de supprimer certaines dispositions déjà redondant dans les sections deux ou trois pour les intégrer dans la section IV qui est plus complète puisqu'elle concerne les différents types de transport lourd, donc c'est un avis défavorable.-- Merci donc je mais aux voix l'amendement 61 du gouvernement avec un avis défavorable de la commission qui est pour.-- Qui est contre.-- Qui s'abstient. Il n'est pas adopté l'amendement 53 je faire monsieur le président, Monsieur le Ministre, chers collègues, la directive. Eurovignette dites Eurovignette révisée prévoit la possibilité d'introduire une redevance de congestion. Sur les 30 tronçons routiers qui sont régulièrement saturés pendant évidemment les périodes habituelles de congestion cette redevance étant facultative. Le gouvernement dans son projet a pris propose de ne pas la transposer. Il nous semble au contraire que pour lutter efficacement contre la congestion et la pollution atmosphérique créée par la circulation se laisser la possibilité de mettre en place cette redevance paraît logique. L'idée de l'amendement et donc d'élargir le Champ de transposition de la directive.-- Il me suis rapporteur.-- C'est monsieur le président, Monsieur le Ministre, chers collègues, la vie, cet amendement est défavorable pour 2 raisons. Il conduit. Vous l'avez rappelé, élargir le Champ d'application de la transposition véhicules légers et pas seulement aux véhicules lourds, l'article sept qu'bis de la directive prévoit en effet qu'une telle redevance de congestion s'applique et de manière non discriminatoire à toutes les catégories de véhicules. Son articulation avec la modulation horaire introduite en commission serait particulièrement complexe. C'est donc une demande de retrait ou un avis défavorable je ministre.--

Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Donc en commission, nous avons adopté un amendement qui permet de faire varier la redevance d'infrastructure afin de réduire la congestion routière ainsi les péages pourront être pourront être modulée en fonction du moment de la journée du type de jour ou de la saison. Nous sommes favorables à cette disposition. Nous considérons que concernant le transport de marchandises, le surplus des recettes pouvant résulter de l'application de ces modulations de péage pourrait être utilisé pour favoriser le développement du report modal ferroviaire et fluvial indispensable pour lutter efficacement contre le changement climatique. Cet amendement propose dès lors d'une part, de rendre possible une augmentation du montant total de recettes liées aux modulations de péage pour des raisons de recevabilité financière il n'a pas été possible de prévoir d'orienter l'éventuel surplus de recettes au soutien du report modal ferroviaire et fluvial moyen de transport efficace pour lutter contre la congestion routière et la pollution atmosphérique. Mais je tiens à souligner que telle est bien l'intention de cet amendement depuis de trop nombreuses années est émis le souhait de mettre en oeuvre un véritable report modal des marchandises transportées sur la route vers le fluvial et ferroviaire en ce qui concerne le fluvial avec 8500 kilomètres de voies Nagui navigable. La France possède le plus long réseau d'Europe qui en compte 38.000 au total mais elle est aussi l'un des plus faibles utilisateurs le transport fluvial de marchandises représente moins de 3% des tonnes kilomètres transportés principalement des matériaux lourds, céréales et BTP en tête, contre 7% en moyenne en Europe. Les voisins belges 12% allemand 15% et surtout hollandais, 43% en font une utilisation beaucoup plus fréquente. C'est un mode de transport qui n'est pas saturé, dont la capacité pourrait pourrait être multiplié par 3 ou 4 et qui permettrait d'acheminer des marchandises au coeur des grandes agglomérations avec la logistique du dernier kilomètre, tout en limitant le recours aux transports routiers terrestre quant au fret ferroviaire de cesser de perdre des parts de marché depuis des décennies. Si nous voulons réussir la massification du transport bas-carbone de marchandises. Nous devons trouver des financements y penser.-- Merci monsieur rapporteur.-- Si monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Cet amendement est contraire aux dispositions de la directive Eurovignette qui prévoit ces articles c'est coauteur bis et 7 obtient 10 que les modulations, non pas pour objet de générer des recettes supplémentaires en août cette situation conduirait simplement augmenter les recettes des exploitants autoroutiers. Donc c'est une demande de retrait ou à défaut un avis défavorable. Merci, monsieur le Ministre. Même avis, il ne s'agirait pas ici de sur-transpositions mais bien comme l'a rappelé monsieur le rapporteur d'une disposition contraire aux textes la directive donc avis défavorable aussi.-- Il est maintenu ou retiré et maintenu donc je mais on voit le 22 avec 2 avis défavorable qui est pour.--

Sorti du fléchage des recettes pour le financement d'infrastructures de transport. Ce nouveau dispositif permet de majorer les péages jusqu'à 50% alors qu'il se limite aujourd'hui à 25. L'étude d'impact à considérer que ce sur péage pourraient être mises en place lorsque des opérations seront identifiés. Pourquoi alors à tendre pourquoi être moins 10 ans alors qu'on peut avoir un dispositif transposer la, la commission d'orientation des infrastructures dont nous sommes tous suspendus à la publication du rapport ne va pas pour autant inventer de l'argent. Il nous faut trouver de nouvelles sources de recettes pérennes destiné à accroître la part du fluvial, celle des mobilités actives encore trop marginal en plus les indispensables projets de régénération une modernisation du réseau ferroviaire. Cet amendement montrerai peut être le chemin. Merci monsieur le rapporteur. Merci monsieur le président, de même que pour l'article 53, cet amendement sont particulièrement complexe à mettre en oeuvre et articulé avec la possibilité de modulation horaire introduite par la commission. Donc c'est une demande de retrait ou à défaut un avis défavorable. Merci, monsieur le Ministre. Même avis monsieur le président. Merci. Il est maintenu. Se faire Nick oui ah les je mais au voile 54 avec 2 avis défavorable qui est pour. Qui est contre qui s'abstient. Il n'est pas adopté 2 amendements en discussion commune de 60 du gouvernement, Monsieur le Ministre.-- Oui, monsieur le président, il s'agit d'un amendement de suppression. L'idéal, elle n'à 19 qui est relatif à l'entrée en vigueur de l'article L 119 tiré 12 du code de la voirie routière. Donc, l'amendement de de modification de cet article du code de voirie routière adopté par la commission là aussi nous semble superflu superflu et pouvant nuire à la compréhension de l'application de la redevance pour co-externes qui est prévu par la directive et donc nous avons lancé plusieurs consultations qui seront soumises à directive Eurovignette. Et la proposition du gouvernement vise à Roche a modifié pour éviter une ambiguïté sur l'application de cette modulation CO2 et des redevances additionnel en attendant le résultat de ces opérations de consultation. Merci de 52 Monsieur.-- M. esprit. Un amendement qui vise, lui a avancé la date d'entrée en vigueur qui a été reculé, par la commission du Sénat à 2024. Merci monsieur le rapporteur.-- Merci Monsieur le Président. Donc ces amendements revienne sur un accord de la commission qui a au contraire estimé que cette prévision relatives à la date d'entrée en vigueur était nécessaire. La directive prévoit que prévoit par ailleurs que la redevance pourquoi externes lié à la pollution atmosphérique due au trafic s'applique de façon obligatoire à compter de mars 2026. Avancée. L'entrée en vigueur de cette obligation conduirait donc il y a une sur-transposition de la directive. En outre, l'application de cette redevance, à partir de 2026, n'empêche pas la mise en oeuvre des dispositions de modulation en fonction du CO2 dès 2022. Elle sera simplement mises en Oeuvres de façon différée afin de permettre aux transporteurs de renouveler leur flotte en vue de cette échéance, ce sera donc un avis défavorable.

Merci, monsieur le Président, j'aimerais faire une petite explication de vote sur l'article de 26 puisque nous allons voter contre cet article. Là on n'avait pas terminé parce qu'il y un amendement. Excusez-moi.

Merci, monsieur le Président, donc nous allons voter contre, l'article 26, cet article nous a interpellés, puisqu'on y voit apparaître une nouvelle redevance sur les transports routiers, payé par les automobilistes et les transporteurs de marchandises. Une fois de plus ce sont les usagers de la route qui sont stigmatisés, à défaut de pouvoir être les usagers d'autres choses, il y a évidemment un enjeu à soutenir la transition des mobilités. Il faut décarboner nos modes de transport qui représente aujourd'hui 30% de nos émissions de CO2 quasi uniquement du fait du transport routier. La logique de sanctionner par une redevance supplémentaire. Celles et ceux qui seraient responsables de cette pollution a du sens, sauf qu'il s'agit là d'un choix par défaut parce que le transport de marchandises par le fret ferroviaire est trop insuffisamment développée et parce que le transport de voyageurs va être développé, mais on ne sait pas quand c'est pour bientôt. Enfin c'est pas pour tout de suite quand même. Avec cette redevance supplémentaire. Il y a la même logique que dans le déploiement des ZFE les zones à faibles émissions qui sont une bonne idée pour améliorer la qualité de l'air mais qui dans les faits condamne toutes celles et tous ceux qui n'ont pas la possibilité de changer leur véhicule à rester chez eux, je pense notamment aux aux aides à domicile et à d'autres salariés également. Avec cette redevance. Les familles continueront de prendre l'autoroute pour partir en vacances en payant plus cher les colis de Noël continueront d'être acheminés par la route et coûteront plus cher la pollution continuera d'exister de toujours nous coûter cher cher en matière de santé et les profits des gestionnaires d'autoroutes oui continueront d'atteindre des records. Pendant que les trains plus économique et écologique resteront OK donc nous allons voter contre cet article, je vous remercie.

qui a pour objectif donc d'adapter le code des transports pour tenir compte des compétences dévolues à l'Autorité de régulation des transports, en matière de système européen de télépéage. Merci. Le 34 Monsieur Lefebvre. Oui c'est le même amendement il a été très bien défendu par Monsieur Beulin. À l'instant. Merci monsieur le rapporteur. Si Monsieur le Président. l'ART lorsqu'elle est saisie dans sa mission de conciliation entre les percepteurs de péages et les prestataires du service européen de télépéage et demander toute information percepteur des péages. Aux prestataires. aux prestataires de service européen de télépéage à toute personne en activité est liée à la prestation du service européen de télépéage. La question de la nécessité de prévoir une nouvelle disposition à portée générale en la matière se pose donc c'est pourquoi je sollicite l'avis du gouvernement sur cet amendement. Merci, monsieur le Ministre.---- Merci, monsieur le Président, j'ai ressenti une forme de réticences sur cet amendement dans le la position même si elle demande un éclairage du gouvernement. Monsieur le rapporteur. Je la partage. Si c'était le sens en effet de votre analyse parce que nous serions sans doute sur la forme. Monsieur le sénateur blanc dans un cavalier législatif puisque nous serions étranger au Champ de transposition de la directive, même si sur le fond, l'extension de prérogatives prévues n'est pas forcément une mauvaise chose mais nous vous demanderions de retirer les amendements qui sont ainsi déposé.-- Merci Monsieur Beulin. Il est retiré. Il est retiré. Monsieur Lefebvre. Aussi 2 amendements sont retirés ne passe nous au vote sur l'article 26 Bis qui est pour.-- Qui est contre qui s'abstient il est adopté. Même vote pour le 27.

Oui, merci Monsieur le Président. Cet amendement a pour obliger d'appliquer aux services urbains sur urbains et régionaux. L'article 8 du règlement relatif à l'obligation de fournir des informations sur l'interruption des services à l'article 30 relatifs à l'information des voyageurs sur leurs droits. Le présent amendement prévoit aussi, conformément à la demande des associations représentatives des usagers d'appliquer aux services urbains et suburbains et régionaux au même titre qu'au service à longue distance. L'article 30 qui impose l'information des voyageurs sur leurs droits et obligations lorsqu'ils achètent des billets de transport ferroviaire ainsi qu'en gare à bord des trains et sur les sites internet des entreprises de ferroviaire et des gestionnaires des gares. Ces informations devront notamment être fournis dans des formats accessibles à tous qu'on a tous conformément à la réglementation applicable, notamment en cas d'annulation de correspondance manquée ou de retard important lors de la vente de billets est envisageable de déterminer les conditions d'assistance aux personnes handicapées et à mobilité réduite en complément en complétant le décret numéro 2021. 1124, pris en application de l'article L. 1115 tiré 9 du code des transports dans l'objectif d'assurer une application cohérente à tous les services ferroviaires urbains et sur Burda qu'ils soient exploités ou non par les entreprises. Dotée d'une licence d'entreprise ferroviaire. Néanmoins, il est essentiel que le décret cité soient publiés avant la date d'entrée en vigueur du règlement européen soit le 7 juin 2023 et que sa rédaction se fasse bien, en concertation avec les associations représentatives. Je vous remercie. Oui il est défendu pas de difficulté simplement. Un message pour le gouvernement. Il est très bien qu'on est noté dans la loi que le décret sera pris après avis du CNCPH. Rappelons que c'est déjà dans la loi de 2005, c'est un principe général.-- Merci de 46 Madame Préville. Oui il a été très bien défendu. Je voudrais juste rajouter comme mes collègues que j'avais un amendement un petit peu différent que ai j'ai rectifié pour le rendre identiques et que nous serons très vigilants sur le contenu du décret.-- Merci de 57. Monsieur.-- Il a été bien défendu. Donc il semble indispensable de retirer certaines des exemptions. Prévues par ce projet pour les services ferroviaires suburbains et régionaux. Certaines dispositions du règlement sur les droits et obligations des voyageurs fait voir. Merci de 77 du gouvernement, monsieur le ministre, il a été défendu.-- Allez, si vous le permettez, et en effet. Je, je partage l'objet des amendements qui ont été présentés. vous propose aurions puisque le texte du gouvernement dans cet amendement est sensiblement destiné aux mêmes objectifs, c'est-à-dire supprimer un certain nombre de dérogations. En effet, je prends le point sur la nécessité de suivre l'application précise par décret. Nous avons eu un échange informel. Avec le CNCPH ces derniers jours que nous allions plus loin dans la non prise en compte de dérogations qui me semble excessif par rapport au texte initial déposé par le gouvernement. Donc je crois que l'amendement 77 que je présente au nom du gouvernement répond aux préoccupations qui ont été exprimées dans les quatre amendements précédents et donc si. Vous en êtes d'accord, je vous demanderai de bien vouloir les retirer au profit de cet amendement 77 en prenant en compte votre demande de vigilance sur les textes réglementaires qui suivront. On a eu du tout. Merci. Sont ils sont identiques. Hein. Monsieur le Ministre. Donc. Alors le 74, madame pour Oui, merci Monsieur le Président. Notre chère collègue notre amendement vise à rétablir la rédaction initiale du texte qui rendait possible les indemnisations le remboursement et l'assistance aux voyageurs dès 2023 la commission de développement durable a repoussé repoussé ce délai de mise en oeuvre à notre. Grand étonnement, comme si la gronde, comme si la colère des usagers des transports en voie de privatisation ne s'entendaient pas suffisamment les suppressions de trains, des retards, les difficultés du quotidien ne rendent pas service au ferroviaire qui a besoin d'un investissement d'ampleur pour redevenir un modèle de ponctualité, de fluidifier fluidité. La plupart des usagers, se retrouvent aujourd'hui à prendre le train par contrainte, davantage que par l'aspect pratique écologique et économique que le transport ferroviaire devrait incarner. Il faut entendre les usagers et il faut répondre à leurs attentes.-- Merci, monsieur le Président donc les amendements 30 rectifié terre 43 rectifié terre 46 rectifié 57 rectifié 77 donc pour répondre à la question du ministre ont été. Mis sur la même rédaction que le gouvernement et je remercie les collègues qui sont prêtés au jeu donc de modifier pour le rendre identiques donc ils permettent d'améliorer l'information des voyageurs ferroviaires en cas d'interruption du service a été rappelé. D'autre part la définition par décret des modalités d'assistance aux personnes handicapées ou à mobilité réduite à un décret pour ce qui concerne les services urbains et suburbains permettra sans doute un renforcement de leurs droits, donc c'est un avis favorable à ces amendements donc le 30 rectifié terre qui entre actualité à 46 rectifié 57 rectifié et le numéro 77. Et donc l'amendement numéro 74 revient quant à lui sur une évolution introduite en commission en rétablissant le texte initial sur ce point, cet amendement pour à la fois conduire à des situations de rupture d'égalité entre différentes catégories de voyageurs ferroviaires et entraver le bon déroulement de l'ouverture à la concurrence, donc c'est un avis défavorable. Merci, monsieur le Ministre.-- Pardon, monsieur le président. Je n'étais pas à 100% à jour. Merci aux sénateurs qui ont proposé sénatrice qui ont proposé des amendements les avoir adapté. Pour qu'ils soient conformes en effet totalement identique à la rédaction de l'amendement 77 donc j'aimais le même avis de soutien à l'ensemble de ces amendements. Quant aux 74 même avis que le rapporteur, il nous semblerait que l'effet souhaité soit pas tout à fait atteint par la rédaction qui irait plus loin et pourrait créer des discussions difficultés pardon d'application de date d'entrée en vigueur. Monsieur le Ministre donc je mets les 5 amendements identiques aux voix le 30 43 46 57 77 qui est pour.-- Qui est contre. Qui s'abstient. Ils sont adoptés. Et il faut tomber donc. Le 74.-- Le 55 Monsieur faire Nick. Oui, monsieur le président, Monsieur le mini chers collègues donc les entreprises ferroviaires doivent dans la mesure du possible, faciliter la combinaison de trajet à vélo avec des trajets ferroviaires. à la popularité croissante des déplacements à vélo le chiffre vient d'ailleurs de tomber. L'utilisation du vélo a encore progressé de 11% pour les 3 premiers trimestres 2022. Au regard des mêmes trimestres pour 2021 et donc c'est bien l'objet du règlement que l'on transpose aujourd'hui que notamment la place du vélo dans le ferroviaire, on avait effectué en France un progrès très important. Grâce à la l'homme en fixant un nombre minimal d'emplacements vélo dans l'été j'avais été T TER au niveau national. Mais vous vous souvenez peut-être la loi trois des s à modifier ce régime pourtant tout nouvellement mise en place en donnant compétence à chaque région pour fixer son propre seuil minimal dans les TER. Cette proposition était régressive ça pour de voir l'ambition du décret revu à la baisse cet amendement vise donc à renforcer la transposition de l'article 6 du règlement Réenclencher dans le bon sens. Définit lorsqu'elle comment du matériel roulant, 9 ans, un nombre adéquat d'emplacement pour bicyclette. Pour autant, le code des transports sont d'ores et déjà prévoir des obligations analogue. Je m'interroge donc sur la nécessité d'introduire cette précision supplémentaire. C'est donc un avis de sagesse. Oui, monsieur le président, pour les raisons qu'a indiqué monsieur le rapporteur, tout en donnant un avis de sagesse, il nous semble que le cadre prévu par la loi d'orientation des mobilités permet d'aller dans le sens que le sénateur faire niquer évoque dans son amendement que nous avons donc les dispositions nécessaires pour le cas échéant, aller plus loin. S'agissant des services urbains et donc je, je vais mettre un avis défavorable à cet amendement. Merci, monsieur le Ministre dont je mais on voit le 55 avec un avis de sagesse de la commission un avis défavorable du gouvernement qui est pour.-- Qui s'abstient. Qui s'abstient. Il n'est pas adopté, je mais aux voix l'article 28 qui est pour l'article 28.-- Qui est contre.--

Oui, merci Monsieur. Le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Je souhaitais rapidement intervenir sur cet article pour émettre quelques réserves et des questionnements sur le bien-fondé des décisions prises ici en effet, cet article pour se mettre en conformité avec la réglementation européenne, confie la gestion des aides à l'installation des jeunes agriculteurs, la fameuse DJIA aux conseils régionaux et il est important que cette régionalisation ne crée pas des inégalités de traitement et des distorsions entre les agriculteurs avec des régions et nous et nous savons bien. Qu'ils font des choix politiques parfois très différents et les politiques publiques en matière d'agriculture n'y échappe malheureusement pas le gouvernement le reconnaît. Même à demi-mot dans son amendement numéro 76 en m'indiquant si l'autorité de gestion régionale déploie cette possibilité à propos de l'acquisition des compétences en cours d'installation, la réalisation d'un bilan annuel de la politique d'installation par région sera ainsi particulièrement utile pour constater des éventuelles des éventuels concernant les conditions minimales de formation pour bénéficier de la DGA. Nous sommes particulièrement étonné de la position du gouvernement l'ajout réalisé en commission par le rapporteur reprend exactement les termes de l'Arctique à 330 tirer 1 du code rural en vigueur qui conditionne actuellement la DGA et aujourd'hui il ne semble pas qu'il y a des problèmes d'attribution de la DGA sur nos territoires. Au contraire, nous considérons que les aides agricoles doivent bénéficier aux agriculteurs avec un projet viable et des compétences liées, Il semble donc aujourd'hui délicat de considérer que pour bénéficier là de la DGA il faudrait être moins disant ans que la législation actuelle. Toutefois, en l'absence d'éclaircissement du gouvernement sur ses intentions, nous nous abstiendrons sur les différents à un moment sur ce sujet.-- Merci. Nous passons à l'amendement 50 Monsieur Oui, monsieur le président, Monsieur le Ministre. Cet amendement a un caractère sérieusement important dans le sens où il permet parce que c'est un amendement de coordination

Cette application de coordination. Eh bien tout simplement la la la loi Dadu viendrait déformées ou annuler. Ce que nous avons voté l'année dernière à l'intérieur de la loi assurance-récolte.-- Si cher collègue de cool. La commission a donné un avis favorable. Oui. Avis favorable, Monsieur. Parce que c'était. C'était un amendement. C'est plus mon amendement, c'est l'amendement de la commission, monsieur le président. D'accord très bien. Monsieur le. Mais. Oui, monsieur le président. Je suis au nom du gouvernement favorable à cet amendement, sous réserve que l'on puisse adopter le suivant. Ou celui qui sera présenté juste après avec 58 rectifié le 76 du gouvernement dont je pourrais présenter les précisions puisque c'est l'ensemble de ce dispositif qui nous semblerait pertinent.-- Donc. Favorable avec réserve. Mais je le mets quand même aux voix l'amendement 50 de la commission, même s'il était du rapporteur à titre personnel mais enfin bon. C'est c'est l'amendement la commission avec un avis favorable sous réserve du gouvernement qui est pour.-- Qui est contre qui s'abstient il est adopté 2 amendements identiques, le 58. Président Gontard.-- Oui, merci Monsieur le Président. Cet amendement vise à supprimer l'obligation de détention d'une capacité professionnelle. Pour l'accès aux aides à l'installation agricole introduite en commission des affaires économiques. En effet, cette mesure est bien plus restrictif que le droit européen et entre en contradiction avec les objectifs de renouvellement des générations de création d'emplois en agriculture et de souveraineté alimentaire. Aujourd'hui, nous le savons et cela sera l'objet de débats dans le cas de la future loi d'orientation agricole ne devons installer massivement des nouveaux agriculteurs dans 10 ans, 48% des chefs d'exploitation auront un âge de la retraite et la France vient de perdre 100.000 exploitations sur les 10 dernières années, soit une baisse de 21%. Le défi est donc de taille pour permettre la transmission des fermes et faire en sorte que les nouveaux installés nombreux mettent en oeuvre des projets viables sur les territoires répondant aux enjeux de la transition écologique et aux attentes des consommateurs. Dans ce contexte, les installations agricoles se pratique de moins en moins dans un schéma de reprise de la ferme familiale. Après un passage. Enseignement agricole. L'agriculture et c'est une très bonne nouvelle a une diversité de profils notamment issus de reconversion professionnelle. Ces profils diversifiés ne passe pas nécessairement par une formation agricole classique permettant l'obtention d'une capacité agricole. Cela ne veut pas dire pour autant qu'ils n'ont pas les compétences nécessaires à la conduite d'un projet viable à la fois sur le plan technique et économique, il mobilise en effet des compétences acquises dans leur présente activité en équerre d'autres via une multitude de circuit en effet pour certains systèmes de production malgré des efforts de la part des établissements agricoles encore trop peu de formations sont proposées et c'est notamment le cas pour des formations en bio ou avec la transformation à la ferme. Des porteurs de projets se forment ainsi via des stages du salariat agricole le Fonds vivez les espaces test ou encore des dispositifs comme les coopératives d'installation en agriculture paysanne et les écoles paysanne le parcours de demande d'aide à l'installation comporte de multiples garde-fous qui permettent de valider ces expériences et de s'assurer du sérieux du projet du candidat, il est donc essentiel de laisser la possibilité à une diversité de parcours de talents et de compétences de venir créer des emplois de la valeur ajoutée et de la résilience pour nos territoires ruraux merci. Oui pour le présenter. Un mot, puisqu'il est en effet identique il il vise pardon à maintenir le cadre actuel en matière d'exigence de formation minimale pour des raisons de rentrer en vigueur du PSN qui ne s'oppose pas à ce que l'on garde de ce cadre minimal. Nous avons besoin d'adopter rapidement puisqu'une fois que le PSN ne sera pleinement en vigueur. On ne peut plus modifier le droit national de la même façon, donc c'est pour cette raison que le gouvernement a présenté un amendement qui vise le même objet, qui a la même rédaction. demande de ces deux amendements qui sont devenues identiques par mutation de l'amendement du groupe écologique qui n'étaient pas identiques au départ où vous demandiez une expérience professionnelle qui était acquise dans la rédaction dit que cette expérience, cette capacité professionnelle était acquise, a été ramené sans modification d'ailleurs du motif à la réalité de l'amendement du gouvernement, c'est-à-dire la suppression totale de ce que nous avions donné. je vous rappelle une chose, Monsieur le Ministre, c'est que. Votre gouvernement, comme beaucoup d'autres auparavant. Ont demandé sans cesse aux agriculteurs. Une multitude d'injonction une multitude, une multitude de règles une multitude de normes. Et vous voudriez aujourd'hui nous faire croire que au préalable pour pouvoir être agriculteur, il n'y a absolument plus besoin ni de capacité professionnelle ni de formation.-- Eh bien c'est exactement ce que je demande, c'est-à-dire que ce qui est dans le PSN.-- C'est que vous demandez à ce qu'un agriculteur. Une fois son parcours accompli est une forme de capacité professionnelle. Moi ce que je dis, c'est que cette capacité professionnelle a minima. Il faut qu'il ait au préalable à son installation

Qu'qui soit une formation professionnelle une capacité professionnelle ou une formation scolaire et si ça n'est pas totalement le cas qui puisse arriver au niveau mais qui est un minimum fixé d'ailleurs je fixe pas ce minimum. Je dis tout simplement, il faut un minimum qui soit fixée au gouvernement la possibilité dans le PSN dans la modification qui est l'article 9 du PSN la modification nécessaire. Donc vous avez tout lieu de pouvoir faire j'arrive absolument pas à comprendre pour tous ceux qui regarderont ces débats comment on puisse être aussi.-- Paradoxal sur les demandes qu'on fait aux agriculteurs et de l'autre côté, être capable de leur dire non vous avez pas besoin de vous former. Tout va bien.-- Donc la vie, c'est quoi. Donc c'est un avis défavorable pour les 2 amendements, puisqu'ils sont identiques. Merci. Donc je mais on voit les 2 amendements identiques 58 76 avec dont celui du gouvernement, avec un avis défavorable de la commission qui est pour.-- Qui est contre.-- Qui s'abstient. Ils ne sont pas adopté l'amendement 64 du gouvernement, Monsieur le Ministre.-- Merci Monsieur le Président c'est un amendement qui vise à assurer dans les meilleures conditions possibles la bascule aux autorités de gestion régionale de la gestion des aides à l'installation, la dotation jeunes agriculteurs et cet amendement a été travaillé par le ministère de l'agriculture de la souveraineté alimentaire en concertation étroite avec les régions, je crois qu'il ne pose à cet égard. Pas de difficultés. Merci monsieur le rapporteur.-- À l'inverse de celui qu'on vient de d'écarter le bon sens veut que pour cet amendement la vie soit favorable.-- Merci donc je mais au voit le 64 avec un avis favorable de la commission qui est pour.--

Oui on sera, je le dis par anticipation favorable au sous-amendement présenté par Monsieur du plomb, mais l'amendement qui est présenté par le gouvernement a-t-il principal vise à mettre en cohérence le Champ de l'habilitation qui est donné au directeur général de FranceAgriMer d'édicter un certain nombre de dispositions réglementaires avec le chant de spécialité, l'intervention de cet établissement, c'est une mise en cohérence qui je pense est importante pour ses missions. Merci le sous-amendement 83 monsieur le rapporteur. Mais monsieur le président, Monsieur le Ministre cette ce sous-amendement est relativement simple, dans la rédaction on arrive à un pléonasme comme monter en haut descendre en bas puisqu'on dit deux fois l'aide aux personnes les plus démunies. Donc cet amendement rédactionnel vise à supprimer ce pléonasme. Et donc a enlevé dans la partie du goût de l'amendement du gouvernement la partie sur la mise en oeuvre de l'aide aux personnes les plus démunies.-- la vie est favorable pour suivi du gouvernement à condition sous-amendement soit adopté. J'ai bien compris donc le sous-amendement 83 je le mais on voit celui de la Commission avec un avis favorable du gouvernement qui est pour.-- Qui est contre qui s'abstient il est adopté, je mais aux voix l'amendement 65 ainsi sous-amendé avec un avis favorable de la commission qui est pour. Qui elle compte qui s'abstient-il être adopté je mets aux voix l'article 30 qui est pour. Qui est contre qui s'abstient il est adopté, je mets aux voix l'article 31 qui est pour qui est compte qui s'abstient-il être adopté. Je vais mettre aux voix l'ensemble du projet de loi d'adaptation au droit de l'Union européenne. Qui est pour, pardon madame Meunier, il y avait une explication de vote oui. Et il m'a amené. Merci monsieur le président. Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Le groupe socialiste votera. Parce que, que nous sommes des européennes et des européens convaincus. Par contre, je redis, les craintes, les inquiétudes. Notamment dans le Champ social parce qu'en ce qui concerne l'accessibilité et je je vous redis monsieur le ministre que pour nous faire l'écho et le porte-parole des associations oeuvrant dans auprès des personnes handicapées. Il ne faut absolument que le gouvernement maintienne le lien avec ses représentants de personnes concernées pour que ce ne soient pas les oubliés des différentes sur ordonnance que vous saurez prendre dans ce domaine. Merci. Nous avons un texte initial qui je pense mériter et la discussion au Sénat a permis, y compris avec des amendements gouvernementaux mais beaucoup issus des différents bancs du Sénat d'de d'être de renforcer encore la protection que permet ce texte sur les droits des personnes en situation de handicap dans nos transports. Je crois que nous étions allé trop loin dans l'activation de l'instinct de dérogations. Et je crois dans la suite de la discussion parlementaire ne pourront aussi regarder en lien notamment avec le CNCPH et des associations. J'ai reçu Monsieur bon il y a encore quelques jours pour ajuster le texte sans précipitation mais encore au cours de la navette parlementaire dans le sens que vous décrivez et ensuite dans la prise d'un certain nombre de textes réglementaires évidemment que vous suivrez avec attention mais je m'engage à ce que nous y allions plus loin que ce qui est aujourd'hui prévue dans le texte même amendé par le Sénat.-- Merci, monsieur le Ministre donc je mais aux voix l'ensemble du projet de loi portant diverses ils. Opposition d'adaptation au droit de l'Union européenne qui est pour.-- Qui est contre.-- Qui s'abstient.-- Le projet de loi est adopté. Mes chers collègues, je vais lever la séance prochaine séance mercredi 14 décembre à 15h pour les questions d'actualité au gouvernement. La séance est levée.